Il suffit pour s’en persuader de s’arrêter sur quelques chiffres : 7 %, c’est la prévision de déficit public qui nous était promise pour 2025 si nous ne faisions rien pour corriger la trajectoire de la déconfiture budgétaire ; dix jours, c’est le retard pris pour le dépôt du projet de loi

en donnant un budget à la France, nous commençons à rassurer les Français, en démontrant notre volonté et notre capacité de faire face à la dégradation vertigineuse de nos comptes publics depuis 2023. C’était essentiel. Le déficit public devrait se redresser en 2025, pour atteindre 5,4 % du PIB. Cela n’a rien de glorieux, nous le savons bien, mais cela marque un coup d’arrêt à l’effondrement budgétaire, et j’y vois les prémices d’un indispensable redressement.

réponse à ceux qui prétendent faussement que l’État n’est pas au rendez vous. Cela m’amène à ma conclusion : non, un bon budget pour un ministère n’est pas par nature un budget qui augmente ! La France, les Français, les gouvernants et les parlementaires que nous sommes doivent changer de culture.

L’épargne des Français est pléthorique. Sachons donc la mobiliser pour financer les défis qui nous attendent dans ce monde en pleine transformation. Tel un athlète, l’État doit retrouver son poids de forme, se muscler pour être plus affûté. Alors

voie vers cet objectif. Aussi, merci à vous, et poursuivons le travail ! Il n’y a pas une seconde à perdre pour notre France. Elle le mérite tant. Sachons être à la hauteur. La Madame la présidente,

En effet, en faisant tomber le Gouvernement, cette censure a privé la France de budget. Depuis lors, nous fonctionnons en service minimum, et les acteurs économiques n’ont pas de visibilité.

Je remercie sincèrement les quatorze membres de la commission mixte paritaire et leurs suppléants, qui se sont réunis la semaine dernière pendant quatorze heures pour aboutir à un texte qui me semble de nature à concilier nos priorités.

Ce texte, préparé par d’autres gouvernements que le nôtre, est un texte de compromis. Il a été construit en premier lieu avec les partis qui nous soutiennent, par ce socle commun dont je veux remercier les représentants et dont nous avons repris de très nombreuses propositions.

d’instruire celui des revenus et des salaires. Nous avons aussi accru nos efforts pour la transformation écologique, le logement, l’éducation nationale et les outre mer.

Qu’elle nous permette d’adopter le budget dont la France a tant besoin ! J’ai donc l’honneur, après nos nombreux débats et les discussions qui ont conduit au vote conclusif de la commission mixte paritaire, de vous présenter le projet de loi de finances pour l’année 2025. La parole

loi de finances, afin de surmonter, ensemble, l’incertitude et l’instabilité budgétaires que nous vivons depuis plusieurs semaines. Sous l’autorité du Premier ministre, et en coopération étroite avec Éric Lombard, j’ai pris deux engagements lors de ma prise de fonctions comme ministre des comptes publics.

lesquels chaque jour passé sans budget aura coûté plus de 100 millions d’euros aux Français, aux acteurs économiques et au pays. Au total, la facture s’élèvera à plus de 12 milliards d’euros. C’est massif c’est de la croissance et de l’argent perdus. L’urgence à agir dans le contexte politique que nous connaissons a nécessité une méthode nouvelle et inédite pour notre pays : trouver un compromis sur l’objet dont découlent toutes les politiques, c’est à dire sur notre budget. notre budget. Après des mois d’instabilité politique, de surenchère et d’irresponsabilité – j’y insiste –, nous avons réussi à trouver un compromis grâce à l’engagement sincère et authentique de toutes les forces politiques qui ont bien voulu y participer. Je veux saluer leurs représentants qui siègent ici, à la chambre haute. Nous avons collectivement prouvé qu’il était possible de discuter, de débattre et de s’opposer sans pour autant bloquer le pays. Cet engagement s’est concrétisé vendredi dernier, après le vote en commission mixte paritaire du projet de loi de finances pour 2025. Le Gouvernement a contribué, à la place constitutionnelle qui est la sienne, à faciliter et à forger ce compromis.

Ces avancées répondent aux enjeux du moment : le contexte international et le retour de la guerre en Europe, la sécurité des Français et la lutte contre l’immigration illégale, la cohésion des territoires et la lutte contre les inégalités et, enfin, le renforcement de nos grands services publics.

d’abord, en tenant l’engagement des lois de programmation militaire, alors que le contexte international exige aujourd’hui plus qu’hier que nous soyons forts et sûrs d’être protégés ensuite, en continuant d’investir pour la sécurité des Français, conformément aux lois de programmation et d’orientation des ministères de l’intérieur et de la justice ; enfin, en redonnant confiance à nos compatriotes ultramarins,

Enfin, vous l’avez dit, monsieur le ministre, nous demandons un effort fiscal exceptionnel aux grandes entreprises et aux ménages aux plus hauts revenus, sans augmenter les impôts des classes moyennes.

C’est un enjeu de crédibilité et de force par rapport aux autres puissances. C’est aussi un engagement moral pour nos enfants et leurs enfants après eux. Le Premier ministre François Bayrou l’a rappelé dans sa déclaration de politique générale devant le Sénat : notre cible est de repasser sous la barre des 3 % de déficit public au plus tard en 2029. Dès cette année, nous réduirons ce déficit à 5,4 % du PIB, contre 6 % en 2024. Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a rappelé que cet effort était accessible, à la condition que nous exécutions strictement et sérieusement ce budget.

toutefois lancer des réformes structurelles pour dépenser mieux et revoir l’organisation de notre action publique, avec les collectivités, dans la sphère sociale et, plus largement, dans toutes nos ramifications administratives.

Je commençais en vous disant que ce budget n’était celui d’aucun parti. Par votre vote, vous pouvez en faire le budget du pays. La France en a besoin. Nous passons

dirai même la marque de fabrique du Sénat. Si le Parlement dans sa totalité pouvait retrouver cette sérénité constructive au profit du redressement des comptes publics, nous en serions tous ravis.

prononcer. Soyons francs : peu importe l’angle avec lequel l’on examine ce budget, peu importent les analyses que l’on peut entendre à propos de la première ou de la seconde partie du texte, certains ont des regrets, quand d’autres y trouvent des avancées.

Nous sommes également déçus de constater le non rétablissement des crédits budgétaires pour la stratégie de normalisation française à hauteur de 4 millions d’euros supplémentaires, mesure défendue par Jean Baptiste Lemoyne. autre regret important a été d’apprendre la suppression de l’augmentation des crédits de 15 millions d’euros par an en faveur de la recherche clinique sur les cancers pédiatriques, que nous avions pourtant obtenue grâce à Xavier Iacovelli. Oui, nous regrettons que ces mesures ne figurent plus dans le compromis qui est présenté aujourd’hui. Mais si nous avons des regrets, nous constatons aussi des avancées, plus exactement des avancées sénatoriales. Je fais bien évidemment allusion à l’effort budgétaire demandé aux collectivités territoriales, qui a été réduit à 2,2 milliards d’euros au lieu des 5 milliards d’euros envisagés par le Gouvernement précédent à l’automne dernier.

Vous en conviendrez donc, mes chers collègues, nous pouvons toutes et tous mettre en avant ce que chaque groupe a pu obtenir, et c’est bien tout le sens d’un compromis. Cette notion est tout sauf taboue dans notre Sénat, une assemblée composée d’une multitude d’anciens maires, donc d’élus locaux, qui connaissent mieux que quiconque ce que le compromis signifie pour avancer. Avancer, c’est bien de cela qu’il s’agit. Oui, notre groupe votera ce budget, car notre pays doit avancer. Le travail de compromis réalisé avec les groupes parlementaires a été considérable, et je tiens ici à le saluer. Le temps est venu d’éclaircir le climat délétère de l’incertitude et d’avancer pour doter notre pays d’un budget et, par la même occasion, d’accorder du temps parlementaire à d’autres thématiques, qui méritent elles aussi notre attention. Mes chers collègues, notre Sénat s’est distingué en examinant l’entièreté de ce budget. Ensemble, distinguons nous encore une fois en faisant preuve de responsabilité. Adoptons ce budget pour la France ! La parole

une chose est sûre : personne n’est satisfait de ce budget, qui était pourtant très attendu des Français, des entreprises et des collectivités locales. La période de disette budgétaire a plongé le pays dans l’expectative et le désarroi. Il devenait donc urgent d’adopter un budget. Face à cette nécessité, le Sénat a joué à plein son rôle de stabilisateur dans un contexte chancelant. Au terme d’un débat budgétaire exigeant, mais frustrant, au moins pour une partie de l’hémicycle, la commission mixte paritaire a choisi de conserver une copie marquée par la dégradation des finances publiques. Disons le, sur le fond, le texte qui ressort de cette CMP

Enfin, les hauts revenus, ainsi que les grandes entreprises, vont prendre une part plus juste dans le redressement des finances publiques pour l’année 2025. On peut s’étonner des lamentations récentes de certains patrons, qui s’étonnent eux mêmes d’être mis à contribution.

méthode de travail à laquelle les radicaux ont toujours été très attachés, celle du dialogue et du compromis. Dans la configuration politique actuelle, cette méthode est la seule qui permettra d’aboutir à une « confiance retrouvée » entre les Français et leurs représentants. La fièvre budgétaire que nous venons de traverser confirme que le Parlement sous la V République ne peut être qu’une chambre d’enregistrement. En matière budgétaire, il doit être associé dès la phase préparatoire, afin de définir avec Bercy et Matignon les grandes orientations. C’est la garantie que les citoyens puissent constater, constater, par la voix de leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, donc consentir à l’impôt. Cette nouvelle pratique des institutions pourrait permettre à la France de retrouver une stabilité et une sérénité dont les Français, les acteurs économiques

le marathon budgétaire inédit que nous avons couru ensemble n’a jamais autant mérité son nom. Il a été jalonné d’épreuves, de discussions nourries depuis le mois d’octobre dernier, mais l’objectif est en passe d’être atteint : l’adoption d’un budget pour 2025. C’est, en soi, une bonne nouvelle, qui qui nous permet d’envisager une forme de stabilité et de garantir le bon fonctionnement de l’État et des services publics, au service de tous. Voilà qui donne un cap aux acteurs économiques et qui est de nature à ramener la confiance.

et que plus d’une quarantaine d’amendements du groupe Union Centriste ont été retenus. Je m’en réjouis au nom de tous. Ces éléments font, je crois, honneur au Parlement. Cette course de fond a donné lieu à de nombreuses heures d’intenses discussions pour aboutir à un compromis constructif. Ce dernier n’est bien sûr pas parfait, chacun a pu le dire, mais ce texte a le mérite d’exister et de donner un cadre budgétaire stable à notre pays pour l’année à venir.

stratégie consistant à réaliser des économies structurelles et faire des choix dans nos politiques et dans l’organisation de l’État. Le niveau d’imposition et de taxation atteint parfois la cote d’alerte

Nous avons veillé à protéger le pouvoir d’achat des ménages, en indexant bien sûr le barème de l’impôt sur l’inflation, ce qui évitera une hausse mécanique de l’imposition des contribuables. De même, un certain nombre de dispositifs ont pu être soit étendus, soit soutenus. Je pense notamment à l’extension du

est équilibré et permet de préserver non seulement les finances publiques, mais aussi le fonctionnement des services publics déconcentrés. Le groupe Union Centriste votera à la quasi unanimité en faveur du texte élaboré par la CMP à l’issue de ce marathon

contre, parce que ce texte reprend, mais en pire, le projet de loi de finances du gouvernement Barnier, gouvernement minoritaire, battu dans les urnes et censuré voilà quelques semaines. Nous voterons contre, parce que nous aurions dû débattre d’un nouveau budget, d’un budget en phase avec les besoins de changement exprimés par les Français. que c’est l’injustice fiscale et sociale qui prime, à la suite d’un triple coup de force. Il s’agit tout d’abord d’un coup de force démocratique, qui maltraite nos institutions.

Cette reprise en main du texte par la majorité sénatoriale s’est poursuivie jusqu’à la commission mixte paritaire, où elle a su organiser une majorité en sa faveur. Et le recours au 49.3, lundi dernier, a définitivement clos le débat.

L’adoption de ce budget est donc un moment de vérité pour la majorité sénatoriale, qui devra assumer sa responsabilité et ses choix politiques face aux élus locaux.

de 12 points d’ici à 2028. On nous dit que l’effort demandé aux collectivités est de 2,2 milliards d’euros, mais, si l’on ajoute la baisse du fonds vert, le gel des dotations, et j’en passe, on sera en fait bien loin du compte ministre, nous savons que ce budget récessif aggravera la crise. Demain, vous viendrez nous expliquer qu’il faudra encore procéder à un nouveau tour de vis… À la fin, que restera t il ? Un pays divisé, vidé de ce qui fait société. Une République remettant en question ses fondamentaux, qui ont pourtant fait sa grandeur. Quel est donc ce gouvernement qui va jusqu’à reprendre les mots et les idées de l’extrême droite et à mettre les collectivités, les services publics, les élus et leurs agents dans des situations impossibles ? Mes chers collègues, j’espère que vous ne jouerez pas les résignés, dans vos territoires, après avoir voté ce PLF. Encore une fois, en matière d’économie et de budget, il n’y a pas de fatalité. Il n’y a que des choix politiques

Pourtant, nous aurions pu imaginer que la période soit au pragmatisme, que l’on cherche à privilégier ce qui marche et ce qui est utile, plutôt que de faire des choix idéologiques, tant notre pays a besoin de stabilité depuis le décrochage

à poursuivre leur politique, dans une dérive idéologique libérale clairement assumée, saupoudrée de régalien, une sorte de libéral conservatisme. Voilà ce qui caractérise en définitive ce budget,

où la République recule, pour des raisons liées soit à la sécurité, soit à la disparition des services publics, soit à l’environnement et au dérèglement climatique. Or, au vu de l’augmentation des températures et au vu des colères populaires rurales ou dans les banlieues, on peut douter de l’efficacité du ruissellement. les comptes de la Nation, force est d’admettre que, durant la phase haute du cycle économique, les rentrées fiscales liées à l’activité ont équilibré le budget.

nous voilà réunis pour achever le long et tumultueux parcours parlementaire du budget pour 2025. Je veux vous dire d’emblée que nous n’attendions pas grand chose de la commission mixte paritaire

Par ailleurs, en CMP, nous avons obtenu une enveloppe de 500 millions d’euros d’investissements dans les trains régionaux et les petites lignes, qui constituent un élément essentiel dans la vie quotidienne. Je me réjouis aussi que nous ayons rétabli l’Agence Bio, une agence essentielle à la transition écologique.

Loin des discours démagogiques sur l’utilité sanitaire d’un dispositif qui ne représente que 0,6 % des soins consommés, nous avons permis de maintenir une sécurité sanitaire pour tous dans notre pays.

générale, nous déplorons les coupes claires dans les diverses missions budgétaires. Par cette austérité, vous cherchez dans les poches de ceux qui n’ont pas créé le problème des solutions qui ne fonctionnent pas

Nous avons entendu les inquiétudes des Françaises et des Français. Nous connaissons les craintes des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, qui attendent d’avoir de la visibilité et de la stabilité pour construire leur propre budget, embaucher, investir et engager leurs projets.

la France a besoin d’un budget. Le Rassemblement national a été, durant cette phase budgétaire, force de propositions concrètes pour nos concitoyens. Si censure il y eut à l’égard du précédent gouvernement, ce fut uniquement pour protéger les entreprises et les ménages d’un alourdissement trop lourd des impôts, qui conduirait inévitablement à la récession.

coupant dans les crédits des agences Théodule inefficaces, en réduisant les dépenses qui ne profitent pas prioritairement aux Français et en s’attaquant au désordre budgétaire. Mais ce budget, nous ne l’aurons pas… En tout cas pas cette fois. À tout le moins, nous avons eu droit à la réhabilitation du terme de submersion…

Alors que la demande populaire unanime est de réduire ce flux et son financement, ce budget ne s’attaque nullement à cette question. Même la droite sénatoriale, trop heureuse de retrouver les ors des ministères, n’a obtenu qu’une baisse dérisoire de l’AME, malgré ses rodomontades, dont nous prédisions qu’elles

Je vais revenir très rapidement sur les griefs de mon groupe pour prendre, ensuite, le temps de parler de l’avenir. Ce budget ressemble finalement à beaucoup d’autres depuis

Pour répondre à l’urgence budgétaire, nous avons fait comme on fait toujours ! Nous avons sorti le livre posé sur l’étagère de la cuisine et répété la même recette avec les mêmes ingrédients : peu de baisses de la dépense publique, réparties en majorité sur les dépenses d’investissement, et une augmentation de la fiscalité à peu près mesurée sur ceux qui produisent de la richesse dans ce pays, c’est à dire les actifs, les classes moyennes et les entreprises. Dans le contexte Dans le contexte que nous connaissons, nous n’avons pas beaucoup d’autres choix que d’accepter ce compromis. Il est le seul qui permette à la France d’avoir un budget et donc au pays de fonctionner.

un nouveau budget. Contrairement aux idées reçues, ce texte n’est pas toujours le meilleur véhicule législatif pour réaliser des économies. Ce sont les réformes qui auront lieu pendant l’année à venir qui nous permettront d’en faire en 2026. Aussi, malgré la situation politique à l’Assemblée nationale, nous devons nous hâter de réformer le pays pour préparer un avenir de sérénité et de prospérité à nos enfants. Les sénateurs de mon groupe n’ont eu de cesse de le répéter lors des débats sur ce budget : l’État ne peut pas et ne ne doit pas tout faire, sinon il fera mal. Nous devons recentrer l’action publique sur la raison d’être de l’État, à savoir ses missions régaliennes. Et puisque le modèle de société auquel les Français sont attachés est celui d’un État stratège, alors celui ci doit faire porter l’essentiel de sa stratégie sur la préparation de leur futur. En cela, l’instruction publique, l’enseignement supérieur, le financement de la transition écologique, la recherche, l’innovation la modernisation de l’action publique sont autant d’investissements stratégiques. En effet, pour réduire la dépense publique tout en modernisant nos administrations, nous allons devoir investir. La proposition du Premier ministre de créer un fonds spécial consacré à la réforme de l’État, financé par la cession d’actifs immobiliers, nous semble une bonne idée. Pour faire des économies, il faut aussi simplifier les normes applicables à tous les acteurs économiques et adopter des réformes de justice économique. Il n’est pas normal, par exemple, que les règles soient aussi différentes pour les salariés du public et du privé, lorsqu’ils occupent des emplois similaires. Mes chers collègues, nous allons

Cela reste vrai, ce PLF est imparfait. Mais comment pourrait il en être autrement ? Préparé par le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal, qui n’introduisait aucun infléchissement dans la trajectoire calamiteuse de nos finances publiques et laissait à notre pays un très lourd héritage budgétaire…

Ce budget est en fait, pour beaucoup, celui du Sénat, qui a tenté de le redresser et de l’améliorer en responsabilité et avec gravité. Il s’agit finalement du budget de la Nation, fruit d’une commission mixte signe de l’affirmation d’un régime parlementaire et d’une méthode nouvelle de dialogue entre le Gouvernement et le Parlement. Ce budget, malgré ses limites, doit permettre à notre économie de retrouver un souffle grâce à la lisibilité qu’il offre. Il est une bouffée d’oxygène pour nos agriculteurs et nos outre mer. Il doit surtout être le début d’un nouveau chemin, pour engager dans la durée la réduction du déficit public par la baisse de la dépense – j’y reviendrai. Je veux donc tout d’abord remercier tous ceux qui permettent à notre pays de disposer d’un budget : vous, madame, messieurs les ministres, par votre écoute et votre action mixte paritaire, Jean François Husson et David Amiel, qui ont su dans le dialogue trouver une voie majoritairement approuvée en commission et acceptable par d’autres ; les équipes de la commission des finances ; et vous tous, mes chers collègues, par les votes que vous allez exprimer ce matin après celui des députés hier. Ce budget répond à cinq exigences fortes. Premièrement, réduire le déficit de nos finances publiques, en le ramenant à 5,4 % en 2025 et en l’inscrivant sur une trajectoire devant nous permettre de renouer avec les 3 % en 2029. C’est essentiel pour réduire enfin le coût de notre dette, la baisse de la dépense. Deuxièmement, répondre aux enjeux du régalien et des lois de programmation de nos armées, du ministère de l’intérieur et de la justice. Troisièmement, refuser toute hausse de fiscalité touchant les classes moyennes, limitée ou non dans le temps. prendre en compte les préoccupations de pouvoir d’achat de nos concitoyens, notamment s’agissant de l’énergie, en ne ramenant pas la fiscalité de l’électricité au delà de son niveau d’avant crise, afin de garantir la baisse effective des tarifs, mais aussi de MaPrimeRénov’,

Les sujets prioritaires dont nous avons à traiter sont de trois ordres : la démographie, l’innovation et la souveraineté. Les conséquences de l’évolution démographique que nous connaissons sont et vont être considérables – elles sont pourtant insuffisamment anticipées sur nos écoles, la prise en charge de la dépendance, les charges de santé, le financement des retraites, l’immigration, l’empreinte carbone, la relation nouvelle au travail, etc. L’innovation autour des transitions – on peut parler du numérique, du dérèglement climatique, des mobilités ou du logement – constitue le deuxième enjeu majeur. est bien sûr la souveraineté, qu’elle soit industrielle, agricole, militaire, sécuritaire, financière ou budgétaire, qui s’impose en clé de voûte de l’ensemble. Voilà quelques balises qui doivent nous conduire vers un retour à la confiance, à l’espoir et au sursaut. Le budget n’est finalement qu’un outil au service d’une vision, d’un projet, pour la France et les Français. Il nous faut commencer à l’esquisser pour ensuite adapter notre maquette budgétaire à un nouveau paradigme. Le contexte actuel ne permet sans doute pas la reconstruction profonde de notre système, mais nous devons, à tout le moins, ouvrir la voie à sa réforme. Nous en avons tant besoin ! Mes chers Mes chers collègues, conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de finances pour 2025 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

est suspendue. La séance est reprise. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses mesures visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole

le législateur a permis la diffusion jusque dans nos champs de notre modèle démocratique, afin que notre politique agricole s’adapte aux réalités des hommes et des territoires. Ce modèle de représentativité, cette représentation des paysans par les paysans eux mêmes, doit être réaffirmé et conforté. Je profite d’ailleurs de cette occasion pour saluer l’engagement essentiel de toutes les candidates et de tous les candidats aux élections des chambres d’agriculture qui se sont achevées vendredi dernier et dont nous attendons les résultats dans la journée. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte répond à un impératif électoral lié au renouvellement des instances des chambres d’agriculture de ne pas empêcher l’élection de nombreux candidats légitimes. Ce risque est induit, vous le savez, par la séparation entre les activités de vente et de conseil qu’a introduite la loi du 30

prochainement – je l’espère – à l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, ce sont les effets pratiques de cette séparation qui nous intéressent. Et ce sont des effets de bord qu’il convient de corriger en urgence. Dans la mesure où, dans les faits, les activités de vente sont conduites notamment par des coopératives, alors que les activités de conseil sont des missions intrinsèques des chambres d’agriculture, le cadre en vigueur empêche un contingent substantiel d’élus, issus des coopératives notamment, de se présenter au bureau de leur chambre d’agriculture. La proposition de loi de la députée Nicole Le Peih répond donc à une situation d’urgence électorale, qu’il n’était pas possible de renvoyer à des discussions futures au regard du contexte électoral dans lequel nous sommes.

Cette dérogation fonctionne. Il est important de la proroger d’ici à ce que la modification plus substantielle des dispositions relatives à la séparation de la vente et du conseil soit votée après examen par l’Assemblée nationale de la proposition de loi dont je viens de parler. Mesdames, messieurs les sénateurs, la présente proposition de loi répond à une urgence que connaissent l’ensemble de nos territoires, y compris l’outre mer. Il était donc impossible d’ignorer la réalité du drame que vivent les Mahorais. le cyclone Chido a complètement dévasté Mayotte, dont les habitants sont aujourd’hui plus préoccupés par l’acheminement de biens de première nécessité et par la réhabilitation des services publics essentiels que par les échéances électorales.

c’est en responsabilité que le Gouvernement a déposé un amendement visant à décaler d’un an la tenue des élections à la chambre d’agriculture de Mayotte, afin que celles ci puissent se dérouler dans des conditions convenables entre la fin de l’année 2025 et le début de l’année

sénateurs, une proposition de loi sur la démocratie en agriculture ne pouvait non plus s’exonérer d’examiner les imperfections qui affectent les élections à la mutualité sociale agricole Outre la resynchronisation de la durée des mandats des délégués des caisses, qui fait l’objet d’un consensus transpartisan, cette proposition de loi permet de revenir sur la limitation du droit de vote qui s’applique aujourd’hui à l’ensemble des personnes qui ne se seraient pas acquittées de leurs cotisations sociales depuis au moins six mois. Cette limitation, je le dis, me pose une difficulté, puisqu’elle porte une double sanction : elle revient à ce que les personnes frappées sur le plan économique et social le soient aussi sur le plan démocratique. C’est donc une injustice que corrige ce texte.

Mesdames, messieurs les sénateurs, dans le cadre de son examen en commission, des amendements sont aussi venus intégrer au texte des dispositions visant à la parité sur les listes électorales présentées pour la MSA. Ces dispositions permettent de poursuivre le combat en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Elles s’inscrivent donc dans le sens de l’histoire. Comme toujours – c’est une règle que je me fixe en politique –, je souhaite que les progrès que nous portons ne s’exonèrent pas des réalités de terrain.

et chacune de participer à la représentativité du monde paysan. C’est également mon ambition que de permettre aux femmes d’être plus nombreuses en agriculture, mieux protégées et ainsi plus visibles. Le projet

ambitieux, mais réaliste. Enfin, le Gouvernement appuie pleinement les dispositions de cette proposition de loi permettant de réaliser des coordinations juridiques s’agissant de l’élection des délégués dans les anciens cantons de la métropole de Lyon. Mesdames, messieurs les sénateurs, les représentants des territoires et gardiens de la démocratie que vous êtes voteront en pleine responsabilité. En effet, nous commettrions une faute lourde en ajoutant à la crise économique et sociale qui traverse le monde agricole une crise démocratique. Je compte donc sur vous pour vous saisir du sujet et offrir à nos paysans une représentation fidèle dans l’ensemble de leurs instances. La parole

nous poursuivons notre marathon législatif agricole pour discuter d’une proposition de loi qui est nettement plus circonscrite que le projet de loi d’orientation, mais qui est tout à fait utile. Cette proposition de loi relative à l’exercice de la démocratie agricole vise non pas à apporter des réponses de fond à certaines problématiques bien connues du monde agricole, mais plutôt à répondre à l’urgence. Déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale par Nicole Le Peih, députée morbihannaise du groupe Ensemble pour la République, elle a été travaillée, si mes informations sont exactes, en lien étroit avec le ministère.

Je le disais à l’instant, ce texte est un texte d’urgence. Cette urgence provient de l’imminence de la mise en place des bureaux des chambres d’agriculture : les élections, qui ont lieu qui ont lieu tous les six ans, sont à peine achevées – les résultats seront proclamés aujourd’hui –, et il faudra reconstituer les bureaux des chambres au plus tard un mois après, c’est à dire le 5 mars

et Franck Menonville – interdit aux associés des coopératives ayant conservé l’activité de vente d’accéder aux instances dirigeantes des chambres, dans la mesure où ces dernières réalisent des activités de conseil aux agriculteurs – c’est même, j’ose le dire, leur raison d’être ! Dans les faits, Dans les faits, cette incompatibilité exclut un large vivier d’agriculteurs engagés qui font vivre notre démocratie agricole et risque de les priver de représentation dans les chambres d’agriculture. Nous avons, au Sénat, alerté de longue date sur l’impasse dans laquelle tout tout cela allait nous plonger et sur le besoin d’aménager la séparation de la vente et du conseil. Les chambres d’agriculture n’ont d’ailleurs pas manqué de nous faire remonter cette question, notamment lors de l’audition en février 2024 devant la commission des affaires économiques. Dans la précipitation, le texte que nous examinons se contente, à l’article 1, de lever l’incompatibilité sans revenir sur la séparation vente conseil en elle même. Autrement dit, c’est un aménagement minimaliste, qui plus est avec l’instauration d’une règle de déport s’agissant des travaux et délibérations concernant l’activité de conseil. Chacun le constatera, l’ambition est très éloignée de ce que le Sénat a voté il y a peu dans le cadre de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur… Pour autant, il va de soi que cet article 1 est nécessaire pour éviter une situation de blocage. Il est nécessaire, mais loin d’être suffisant. La Coopération agricole l’a d’ailleurs redit elle même publiquement. Il serait dommage de s’arrêter en si bon chemin. Pour le reste, le texte initial contenait trois articles, les deux autres portant sur divers aménagements des élections à la mutualité sociale agricole l’article 2 tend à supprimer la condition d’être à jour de ses cotisations, qui était bloquante pour participer aux élections, et précise la délimitation de la circonscription de la métropole de Lyon ; l’article 3 tend à réaligner les dates auxquelles auront lieu ces élections, car le covid 19 a tout désorganisé. Autant de mesures techniques, sur lesquelles nous n’avions pas d’objections. Le Gouvernement avait initialement exprimé son souhait que le Sénat adopte ce texte dans les mêmes termes qu’à l’Assemblée nationale, afin de gagner du temps et d’éviter une nouvelle lecture ou tout du moins une commission mixte paritaire. Nous souscrivions à cette intention. Seulement, cinq nouveaux articles ont été ajoutés à l’Assemblée nationale, dont un en particulier nous semblait bloquant. Notre commission a donc adopté un amendement de suppression de notre collègue Franck Menonville.

Si nous sommes, au Sénat, plutôt réservés sur les demandes de rapport, celle ci se révélait particulièrement inopportune. Aussi, c’est d’un texte expurgé de cette demande de rapport que nous allons discuter ce jour, ce qui devrait conduire le Gouvernement à réunir une commission mixte paritaire dès lundi prochain. En la matière, j’ai toute confiance dans le Gouvernement pour aider les parlementaires que nous sommes à respecter l’échéance d’une promulgation au avant le 5 mars d’autant plus qu’au delà de ce désaccord, somme toute mineur, ce texte est largement transpartisan, comme en témoignage d’ailleurs le nombre réduit d’amendements dont nous nous apprêtons à débattre. Certaines mesures ajoutées à l’Assemblée nationale ont, du reste, renforcé la pertinence et l’urgence du texte. Je pense en particulier à l’amendement que Mme Le Peih a déposé afin de reporter les élections des chambres d’agriculture à Mayotte, créant l’article 1 B. Cette disposition avait été jugée irrecevable dans le cadre de l’examen du projet et nous devions donc lui trouver un véhicule législatif adapté. Cette proposition de loi sur la démocratie agricole le permet, qui confirme le caractère d’urgence de ce texte, en attendant des réformes plus substantielles. Songeons que, à Mayotte, et pour ne parler que du secteur agricole, 90 % de la production maraîchère et fruitière a été détruite, que l’élevage a été durement touché et que l’essentiel des bâtiments est endommagé ou détruit. Dans ce contexte terrible pour le département, il paraît très difficile d’envisager la bonne tenue des élections de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture suivant le calendrier électoral initial. La démocratie agricole doit pouvoir s’exprimer dans des conditions minimales de sérénité, qui ne sont malheureusement pas remplies actuellement. La parole

ce texte ne modifiera en rien la gouvernance des chambres d’agriculture, car on ne change pas les règles du jeu pendant le dépouillement d’un scrutin. Ce texte n’a pas non plus pour objet de trancher le débat de fond sur la séparation entre la vente et le conseil en matière de produits phytosanitaires. Non Il prévoit simplement de faciliter le déroulement des prochaines élections au sein des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole, en apportant une solution aux problèmes soulevés par ces deux scrutins.

territoires, en raison de l’impossibilité de cumuler un mandat de président ou de membre du bureau d’une chambre d’agriculture et une fonction exécutive à la tête d’une entité chargée de la vente de produits phytopharmaceutiques. Encore une fois, ce choix

n’avions pas anticipé le fait que la grande majorité des coopératives agricoles se spécialiseraient dans la vente et la distribution de produits phytopharmaceutiques. De leur côté, les chambres d’agriculture se sont logiquement tournées en grande majorité vers l’activité de conseil. de ces choix l’impossibilité, pour la quasi intégralité des présidents et des administrateurs de coopératives, d’être élus président ou membre du bureau d’une chambre d’agriculture. D’après Chambres d’agriculture France, la part des personnes concernées par un cumul se situerait entre 15 % et 20 %, mais ce taux s’élèverait à plus de 25 % dans certaines chambres et atteindrait 40 % dans trois d’entre elles : dans les départements de l’Aisne, de l’Eure et de la Moselle. L’implication des coopératives dans les bureaux des chambres leur permet d’avoir une vision partagée sur la transmission des bonnes pratiques et, surtout, sur la diffusion des nouvelles technologies. Leur absence pourrait donc être préjudiciable au développement de certaines expertises.

Néanmoins, malgré l’intérêt que je porte à cette proposition de loi, je regrette que les enjeux de pluralisme et de représentativité n’y soient pas évoqués, au motif, certes, que les élections se déroulent actuellement.

Elle s’inscrit aussi dans une longue série de textes consacrés au secteur agricole, série qui nous oblige à faire preuve de cohérence et à ne pas rendre encore moins lisibles des situations parfois déjà bien complexes. Concrètement, ce texte sur la démocratie agricole prolonge l’aménagement de la séparation entre les activités de conseil et de vente que nous avons adoptée ici même voilà quelques jours.

soulignait en 2023 que cette interdiction de cumul posait des « problèmes techniques et juridiques [pouvant] constituer de véritables points de blocages ». Dans un souci de cohérence et de transparence, les députés ont exigé en contrepartie l’instauration d’une règle de déport, afin d’empêcher les administrateurs membres des exécutifs des chambres d’agriculture de participer aux travaux aux travaux et aux délibérations relatifs à l’activité de conseil en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Les députés ont par ailleurs introduit dans le texte le report d’un an des élections à la chambre d’agriculture de Mayotte. Ce report est parfaitement compréhensible et légitime, eu égard aux circonstances sociales et économiques que connaît l’archipel depuis qu’il a été frappé par le cyclone Chido. La commission des affaires économiques a supprimé, à juste titre, l’article qui prévoyait la demande d’un rapport sur l’opportunité d’adopter un mode de scrutin à la proportionnelle intégrale pour les élections aux chambres d’agriculture. Il n’en demeure pas moins qu’une réflexion sereine et apaisée sur la juste représentativité des chambres d’agriculture aurait tout son sens dans la perspective des élections de 2030.

Il est proposé d’améliorer la représentativité de cette instance en prenant en compte les votes des exploitants qui ne seraient pas à jour de leur cotisation. Cette mesure bienvenue témoigne malheureusement des difficultés de notre tissu agricole. Il aurait été injuste que les exploitants les plus fragiles ne puissent élire leurs représentants dans ces instances. Enfin, le texte permet également d’harmoniser les dates des élections des différentes caisses de la MSA, dont le décalage n’était que la conséquence de la crise sanitaire de la covid 19.

de mesures permettant une meilleure représentativité au sein des instances de gouvernance du monde agricole et de dispositifs s’inscrivant dans le long travail législatif amorcé depuis plusieurs semaines à vos côtés, madame la ministre, pour répondre aux attentes et aux besoins des agriculteurs. Pour toutes ces raisons, le groupe Union Centriste votera cette proposition de loi.

Les élections des membres des chambres d’agriculture, qui précèdent l’élection des bureaux et de la présidence de chaque chambre, viennent de se dérouler. Jusqu’à présent, les dispositions de la loi Égalim de 2018 rendaient compliquée la désignation du bureau des chambres, En effet, cette loi impose une séparation entre les instances qui exercent une mission de conseil et celles qui exercent une mission de vente de produits phytopharmaceutiques. exclut de fait les coopératives agricoles, dont les représentants sont pourtant, en règle générale, issus du monde agricole. Ces personnes seraient donc exclues des bureaux des chambres d’agriculture et du conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. la présente proposition de loi prévoit de permettre aux administrateurs de coopératives agricoles de participer aux bureaux des chambres d’agriculture. Cette possibilité leur sera ouverte ouverte à la condition qu’ils prennent l’engagement de ne pas prendre part aux discussions portant sur l’activité de conseil. Les premiers vice présidents des chambres d’agriculture de région dépourvues de chambre territoriale pourraient entrer dans la composition de Chambres d’agriculture France. La proposition de loi renforce aussi les obligations de publicité des travaux des chambres d’agriculture.

en réduisant progressivement la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête et, d’autre part, de procéder à un décompte des voix à l’échelle du canton. La proposition de loi prévoit également de sécuriser juridiquement les dispositions encadrant l’élection des assemblées générales et des conseils d’administration des MSA.

La séparation de ces activités est motivée par le souci de limiter les recours aux produits phytopharmaceutiques. Mais être candidat à un poste institutionnel

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui portait initialement un titre ambitieux : « Exercice de la démocratie agricole ». Ce titre prometteur laissait espérer une refonte en profondeur de la gouvernance agricole pour une meilleure représentativité de tous les acteurs du secteur. Malheureusement, la proposition de loi qui nous est présentée ne tient pas cette promesse. Elle ne contient que des ajustements à la marge et ne s’attaque pas aux véritables enjeux démocratiques. Le cœur du texte, notamment son article 1, soulève de nombreuses interrogations. Il revient sur la séparation entre la vente et le conseil de produits phytosanitaires, en permettant aux vendeurs, notamment les coopératives agricoles, de siéger dans les chambres d’agriculture. Cette séparation avait pourtant été actée en 2018, dans la loi Égalim, pour éviter les conflits d’intérêts. cette proposition de loi réintroduit ce mélange des genres, sous prétexte qu’on manquerait prétendument de candidats dans certaines régions. Plutôt que d’affaiblir les règles existantes, il eût fallu s’attaquer aux racines du problème la faible attractivité de ces instances pour certains agriculteurs et la nécessité d’un scrutin réellement représentatif. Car c’est bien là le point central : la démocratie agricole ne peut exister sans pluralisme. Aujourd’hui, les chambres d’agriculture sont dominées par un seul syndicat, la FNSEA et ses alliés.

qui favorise la majorité en place et empêche l’émergence d’autres sensibilités. Pourtant, la diversité syndicale existe réellement dans le monde agricole. Elle doit pouvoir s’exprimer à travers un scrutin plus juste, fondé sur la proportionnelle, afin de refléter la pluralité des modèles agricoles et des aspirations des des agriculteurs. Cette absence de pluralisme a des conséquences bien concrètes. Les petits producteurs indépendants, les agriculteurs pratiquant des modèles alternatifs et même les salariés agricoles, pourtant plus nombreux que les exploitants, sont largement sous représentés. Or une chambre d’agriculture doit être un lieu d’échange et de construction collective, non le bastion des tenants d’une seule vision de l’agriculture. Le verrouillage actuel des instances empêche une véritable prise en compte des préoccupations de tous, notamment celles des nouvelles générations d’agriculteurs, qui souhaitent concilier production et respect de l’environnement. Un autre point fondamental est la place des coopératives dans la gouvernance des chambres d’agriculture. Il ne s’agit pas de nier leur rôle dans l’organisation du secteur, mais leur fonction première reste avant tout commerciale. Elles tirent l’essentiel de leurs revenus de la vente d’intrants, notamment de pesticides, et non, hélas ! de la simple collecte des productions agricoles. Dès lors, leur intégration sans contrepoids dans les instances de décision des chambres d’agriculture pose problème. En somme, si cette proposition de loi met en lumière certains dysfonctionnements de la gouvernance agricole, elle n’y apporte pas de solutions concrètes. Pis, en revenant sur la séparation entre la vente et le conseil, elle risque d’aggraver les conflits d’intérêts au sein des chambres d’agriculture. Si nous voulons réellement renforcer la démocratie agricole, il faut aller bien plus loin : réformer le mode de scrutin, garantir un véritable pluralisme, diversifier la composition des instances et assurer une répartition plus équitable des financements. Nous disposons donc de cinq années pour remettre le métier sur l’ouvrage, afin que les prochaines élections des chambres d’agriculture puissent être l’occasion de mieux prendre en compte les attentes de la société et de favoriser une transition agricole en phase avec les enjeux actuels.

Les paysans, et ils sont nombreux, qui déplorent de ne pas se sentir représentés ou d’être mal représentés au sein des instances agricoles devront malheureusement se contenter d’une adaptation, en lieu et place d’une réforme.

Nous ne parlerons donc pas de démocratie agricole, pas plus que de l’épineuse question de la représentativité au sein des chambres d’agriculture. Loin de témoigner de cette – fausse – ambition initiale, induite par un intitulé ronflant, ce texte demeure avant tout technique. Il est censé régler les dysfonctionnements du corps électoral de la MSA, acter le report plus que légitime des élections consulaires à Mayotte, compte tenu de la situation dramatique de l’île depuis le 14 décembre dernier, et proroger le dispositif dérogatoire autorisant le cumul au sein des chambres entre activités de conseil et activités de vente et de distribution de produits phytosanitaires. phytosanitaires. On peut s’interroger sur la pertinence du calendrier : déposé et examiné en quinze jours à l’Assemblée nationale au mois de novembre dernier, ce texte arrive au Sénat en plein renouvellement consulaire.

ou de distribution de pesticides de cumuler ces deux fonctions, sous réserve de ne participer ni aux travaux ni aux délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de ces produits.

La loi Égalim imposait donc aux administrateurs des coopératives, s’ils pouvaient toujours être élus au sein d’une chambre, de ne pas faire partie d’un exécutif. Cette règle de non cumul n’a cependant jamais été appliquée. Dès avril 2019, un processus dérogatoire a été mis en place

de représentation au sein des chambres. Certains considèrent comme une impérieuse nécessité la prolongation de ce dispositif. Nous ne nous y opposerons pas. D’autres en réclament un nouveau, reposant sur la création de certificats d’économies de produits phytosanitaires. Rien ne garantit cependant qu’il serait plus efficace que le dispositif actuel pour aider la France à

Afin de limiter les conflits d’intérêts, cette autorisation de cumul est en effet conditionnée à la pratique du déport, qui interdit à un élu se trouvant en situation de cumul de participer aux travaux et aux délibérations concernant l’activité de conseil. Comme l’a souligné très justement la rapporteure à l’Assemblée nationale, « la règle du déport doit être pleinement appliquée ». Mais de quelle façon ? Il n’existe à ce jour aucune mesure garantissant la bonne application de cette règle. Nous proposerons donc de créer des sanctions en cas de non respect de l’interdiction de participer aux débats. La plupart des autres articles ne nous paraissent pas poser de difficultés majeures. Je reviendrai toutefois sur deux d’entre eux. Nous adhérons aux objectifs de l’article 1 A, introduit par la rapporteure, qui prévoit de renforcer les obligations de publication

L’article 2 prévoit les dispositions relatives aux élections de la MSA, notamment les modalités à mettre en œuvre dans la métropole de Lyon. Nous souhaitons réintroduire dans cet article une disposition qui a été supprimée en séance publique par les députés. Son second alinéa précisait initialement que les personnes n’étant pas à jour de cotisation auprès de la MSA ne pouvaient pas être candidats aux élections de l’instance. S’il ne nous paraît pas indispensable d’être à jour de cotisation pour voter, sachant en outre que les vérifications de mise à jour de cotisation sont des opérations lourdes en termes logistiques, il est pour le moins curieux de ne pas respecter

nous sommes entrés de plain pied dans une séquence agricole particulièrement dense. Je m’en réjouis, tant les sujets sont nombreux et les situations à traiter souvent complexes. Nos agriculteurs ne comprendraient pas que nous n’agissions pas avec célérité, alors que leur activité est sérieusement menacée et que l’avenir des exploitations est incertain. Ces sujets sont essentiels. Et le court texte que nous examinons aujourd’hui, bien qu’il soit de nature technique, a pour objet de résoudre des difficultés très concrètes. La proposition de loi permet de répondre à deux situations d’urgence : les élections à venir au sein des chambres d’agriculture et celles des délégués et des administrateurs de la mutualité sociale agricole.

En revanche, il permet aux associés coopérateurs et membres de coopératives vendant des produits phytopharmaceutiques de participer aux instances dirigeantes des chambres d’agriculture. Qu’ils ne participent pas aux travaux et aux délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est parfaitement compréhensible ; qu’en revanche ils ne puissent pas être membres du bureau ou présider une chambre d’agriculture ne l’est pas. La question de la séparation de la vente et du conseil a été évoquée à de nombreuses reprises ces dernières semaines, notamment lors de l’examen de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. Par ailleurs, comme c’est indiqué dans plusieurs rapports, il nous faudra discuter d’une réforme plus générale, mais tel n’est pas l’objet du texte aujourd’hui. Nous devons à l’Assemblée nationale un apport important : le prolongement d’un an des mandats des membres de la chambre d’agriculture de Mayotte. Cette mesure était indispensable, la situation actuelle, conséquence du cyclone Chido, ne permettant pas d’envisager la tenue des élections.

Dès lors, il était indispensable de réduire ou d’allonger la durée des mandats, afin d’harmoniser autant que possible leurs dates d’échéance. Par ailleurs, cette proposition de loi de bon sens tend, au delà des urgences, à mettre fin à certaines anomalies. Ce texte vise en premier lieu à étendre le droit de vote aux élections de la MSA à l’ensemble des assujettis, y compris à ceux qui sont débiteurs de cotisations réclamées depuis plus de six mois. Ils étaient jusqu’à présent exclus du corps électoral. Cette mesure de simplification est bienvenue, au regard du principe d’égalité du suffrage. Une autre avancée louable pour la MSA mérite d’être signalée : l’article 4 instaure la parité sur les listes électorales des candidats aux élections des délégués cantonaux du deuxième collège. En 2022, quelque 38,6 % de l’ensemble des salariés affiliés au régime agricole étaient des femmes, soit 688 000 femmes. Comme cela a été rappelé à l’Assemblée nationale, nous devons encourager leur participation pour rétablir un équilibre.

Cette première étape peut ainsi rassurer ceux qui s’interrogent sur leur manque de parité ou de transparence. En conclusion, si ce texte prévoit de traiter des difficultés à brève échéance, il ouvre également la réflexion sur d’autres sujets qu’il conviendra d’approfondir dans un second temps et dans un autre cadre, comme la séparation de la vente et du conseil, que nous avons déjà évoquée. Au vu des échanges qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale et en commission des affaires économiques du Sénat, ce texte va dans le bon sens. C’est pourquoi notre groupe soutiendra sans réserve son adoption. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le Sénat est particulièrement mobilisé sur les questions agricoles, ce dont je me réjouis.

la démocratie agricole. Je tiens à saluer le travail de tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce texte. Nos institutions agricoles jouent un rôle essentiel. Dans mon département, la Mayenne, comme ailleurs, les chambres d’agriculture contribuent à structurer l’agriculture locale, à préserver son tissu économique et à assurer la transition des exploitations agricoles face aux défis de demain. puissent continuer de remplir efficacement cette mission, il est essentiel qu’elles bénéficient d’un cadre juridique et démocratique adapté à leurs besoins. Or certaines dispositions législatives récentes ont suscité des inquiétudes, du fait de leurs effets sur la gouvernance des chambres d’agriculture.

L’article 1 permet ainsi d’éviter des restrictions excessives, tout en préservant l’indépendance des conseils donnés aux agriculteurs, notamment en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Je souhaite également saluer la décision de reporter l’élection de la chambre d’agriculture, de pêche et d’aquaculture de Mayotte, en raison des circonstances dramatiques auxquelles l’île fait face. Le vote de

Des associés coopérateurs et des administrateurs de coopératives figurent déjà sur les listes électorales, dans l’espoir que ce texte facilitera leur nomination aux instances dirigeantes dans les délais impartis. Nous devons légiférer rapidement pour garantir le bon fonctionnement et la légitimité de nos instances agricoles. En réponse aux perturbations causées par la crise sanitaire, ce texte permet également d’ajuster la durée des mandats électifs pour les élections de 2025 de la mutualité sociale agricole. Ces mesures sont conformes aux demandes des syndicats agricoles, qui insistent sur l’urgence de les adopter. Il est indispensable de régulariser ces élections pour préserver la stabilité de nos institutions agricoles.

la possibilité de se faire entendre et de participer pleinement à la vie démocratique de cette instance sociale. Cette mesure est essentielle pour préserver l’équité du système électoral et assurer une représentation plus juste de l’ensemble des exploitants, y compris de ceux qui traversent des périodes de fragilité économique – ils sont actuellement nombreux. Au delà de l’accès aux urnes, cette disposition contribue à renforcer l’engagement des agriculteurs dans la gouvernance de leur protection sociale. C’est un pas supplémentaire vers une démocratie agricole plus ouverte, plus représentative et plus protectrice des réalités du monde rural. En somme, ce texte constitue un premier pas, mais il est essentiel de le voir comme une étape vers des solutions durables. Nos agriculteurs, confrontés à des enjeux économiques, environnementaux et sociaux majeurs, ont besoin de structures solides, d’une représentation démocratique renforcée et d’un cadre législatif stable pour accompagner leur développement. Ce texte apporte des ajustements nécessaires, mais il doit s’inscrire dans une réflexion plus large sur l’avenir de notre modèle agricole. Saisissons pleinement cette proposition de loi comme une occasion d’aller plus loin, de poser les bases d’une agriculture plus résiliente, plus compétitive et plus équitable ! Ce n’est qu’ainsi que nous assurerons la pérennité de nos exploitations et le dynamisme de nos territoires ruraux.

nous sommes ici pour examiner une proposition de loi de notre collègue députée Nicole Le Peih. Sous des aspects techniques, ce texte répond à des enjeux essentiels pour notre agriculture, notamment nos chambres d’agriculture. nos chambres d’agriculture. Celles ci, nous le savons, jouent un rôle central dans l’organisation et le développement du monde agricole. Nous devrions connaître le résultat des élections aujourd’hui, et je salue celles et ceux qui se sont engagés. Ces chambres sont à la fois un relais entre l’État et les agriculteurs, un outil d’accompagnement, un espace de dialogue et une force de proposition pour faire évoluer notre modèle agricole en représentant l’ensemble des acteurs de ce milieu

voterons. Ce texte corrige une incohérence issue de la séparation des activités de vente et de conseil pour les produits phytosanitaires. En effet, les administrateurs de coopératives agricoles étaient empêchés de siéger au sein des bureaux des chambres d’agriculture. Il était difficile d’expliquer à un agriculteur qu’un responsable de coopérative, qui connaît son territoire, ses besoins et les réalités de sa profession, ne puisse pas pleinement participer aux décisions des chambres d’agriculture, alors même qu’il en est un acteur clé. En rétablissant cette possibilité, nous permettons à nos chambres d’agriculture de retrouver une gouvernance plus équilibrée et plus représentative. En outre, ce texte introduit une règle de bon sens : l’obligation pour chaque chambre d’agriculture de se doter d’un règlement intérieur. Cela peut sembler une évidence. Pourtant, jusqu’à présent, rien n’imposait aux chambres d’agriculture d’adopter un tel document. Le règlement intérieur est un outil essentiel pour garantir un fonctionnement clair, stable et conforme aux principes démocratiques. Il définit les règles du jeu, encadre la prise de décision et assure une meilleure gouvernance interne. Il s’agit donc d’une mesure qui va dans le sens d’une plus grande transparence et d’un meilleur fonctionnement des chambres d’agriculture. Enfin, ce texte s’inscrit dans l’effort de simplification auquel nous sommes attachés, ici au Sénat, notamment en facilitant la participation des exploitants agricoles aux élections des délégués et administrateurs de la MSA. Actuellement, les

Ensuite, elle complique la constitution des listes électorales de la MSA, en excluant certains exploitants pour des raisons administratives. En levant cette restriction, nous faciliterons la participation des agriculteurs à la gouvernance de leur propre système de protection sociale. protection sociale. Ce texte sécurise également l’organisation des élections des membres de la MSA pour 2025 en harmonisant les dates des différents scrutins. En conclusion, ce texte est utile, pragmatique et attendu. Certes, nous aurions préféré un vote conforme. Certes, la demande de rapport introduite par l’Assemblée nationale à l’article 1 est sûrement superflue. Mais l’essentiel est préservé.

où nos exploitants sont confrontés à des défis majeurs. Ce texte vise à renforcer la représentativité et la transparence des institutions agricoles. Les chambres d’agriculture, qui fêtent leur 101 anniversaire ce mois ci,

Les règles actuelles d’élection aux chambres d’agriculture, notamment depuis la loi Égalim 1, respectent le principe de séparation ferme des activités de vente et de conseil pour les produits phytopharmaceutiques, qui exclut, de fait, les administrateurs de coopératives agricoles. Ce texte propose une solution d’équilibre : sans revenir sur le principe de séparation établi par la loi Égalim 1, il permet aux administrateurs d’être élus aux instances dirigeantes des chambres d’agriculture, mais leur interdit de participer à l’activité de conseil quant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Cette mesure répond aux impératifs d’intégrité, tout en enrichissant le débat démocratique au sein de ces institutions. La MSA, elle, garantit la protection des exploitants, des salariés et de leurs familles en matière de santé, de retraite et de prestations sociales. Pourtant, des rigidités administratives et des contraintes de gouvernance freinent son adaptation aux évolutions du secteur. Cette proposition de loi apporte des solutions concrètes pour moderniser son fonctionnement et mieux accompagner les agriculteurs, dans une période de grande incertitude. Parmi les propositions majeures, l’article 3 du texte prévoit une adaptation du calendrier des mandats des représentants de la MSA. Face à la crise agricole actuelle, il est essentiel de garantir une continuité dans la gouvernance de cette institution. Ainsi, ce texte permettra au ministre de l’agriculture de fixer par arrêté la durée du mandat des délégués cantonaux et des administrateurs de la caisse centrale jusqu’au 31 décembre 2025. telle mesure permettra d’harmoniser les échéances et de mettre en place un calendrier électoral unifié pour l’ensemble des instances de la MSA en 2025, ce qui assurera une meilleure transition dans la gestion des prestations sociales agricoles. autre avancée significative est la suppression d’une disposition contraignante qui empêchait certains exploitants de voter lorsqu’ils avaient plus de six mois règlement de leurs cotisations. Cette barrière administrative nuisait à la représentativité et privait certains agriculteurs de leurs droits démocratiques. Désormais, chaque exploitant, même en difficulté financière, pourra pleinement participer aux décisions qui les concernent. En outre, cette réforme introduit une parité progressive dans les élections internes de la MSA. Dès 2030, les listes de candidats devront alterner hommes et femmes, garantissant ainsi une représentation plus équitable des acteurs du monde agricole. C’est une avancée majeure pour la diversité et la représentativité au sein de cette institution. Ces évolutions sont non pas de simples ajustements techniques, mais de véritables améliorations, pour que la MSA reste une institution efficace et juste, pilier du monde agricole. Ce texte nous engage collectivement à renforcer notre modèle social agricole, à garantir des institutions plus accessibles et plus démocratiques et à soutenir nos agriculteurs dans les défis de demain.

en cas de non respect de cette obligation. En renforçant les garanties d’impartialité, il préserve l’intégrité des missions des chambres d’agriculture et accroît la confiance dans leur fonctionnement. On parle beaucoup de confiance et de transparence : nous devons mettre en œuvre

pour les personnes qui seraient réautorisées à devenir membres du bureau d’une chambre, lors des travaux et délibérations concernant l’activité de conseil et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Je rappelle, au nom du

a pour objet de rendre obligatoire l’adoption d’un règlement intérieur garantissant le pluralisme et la transparence, afin de renforcer la représentation équilibrée des différentes organisations agricoles et d’assurer une traçabilité des délibérations et des décisions prises. Cette mesure s’inscrit dans une démarche de modernisation et de démocratisation des chambres d’agriculture. Son but est de renforcer leur légitimité et leur exemplarité,

séances des chambres d’agriculture ne sont pas publiques, mais que les chambres peuvent décider la publication de leurs procès verbaux. En rendant systématique la publicité des travaux, l’adoption de cet amendement contribuerait à prévenir d’éventuels conflits d’intérêts et à renforcer la transparence du dispositif.

Il nous semble intéressant d’engager une transition vers un scrutin proportionnel pour les élections professionnelles agricoles. Cela renforcerait le pluralisme et la représentativité au sein des chambres d’agriculture.